Républicains. Monsieur le Premier ministre, j'aurais préféré vous souhaiter la bonne année. Je le fais tout de même, mais vous comprendrez que, depuis cette interview du Président de la République, aussi sidérante que désolante, les mots d'Emmanuel Macron sont dans tous les esprits. Ces mots, je ne les prononcerai pas. Je ne les prononcerai pas ici, au Sénat ; je ne les prononcerai pas, parce qu'ils n'ont pas droit de cité dans notre conversation civique. Aucune urgence sanitaire ne justifie des propos d'une telle brutalité, d'une telle indignité. Et Sarkozy alors ? Aucune nécessité épidémique ne légitime qu'un président de la République qu'un président de la République aille jusqu'à dénier à ses propres compatriotes la qualité de concitoyens. Monsieur le Premier ministre, celui qui vous parle est vacciné. J'ai voté- vous le savez -le passe sanitaire. Mes chers collègues, je voterai le passe vaccinal, malgré ces provocations calculées, malgré le piège qui nous est tendu. C'est une honte Monsieur le Premier ministre, je vous interroge : dans une France qui est tellement facturée, morcelée, « archipélisée », pensez-vous qu'il faille en rajouter, encore, en division, en discorde ?

Maire, auriez-vous utilisé ces mots-là, avec ce sens-là ? Telle est ma question.

Oui, nous avons l'impérieuse nécessité- nous le faisons depuis des mois -de faire progresser la vaccination dans ce pays. Vous braquez les non-vaccinés mais, comme vous- je n'en doute pas -, je vais sur le terrain. Vous avez bien voulu faire allusion, cher président Retailleau, à mes anciennes fonctions de maire : quand, comme vous, je me rends très régulièrement dans les services de soins critiques, ce qu'a dit le Président de la République, je l'entends partout. Mais bien sûr que oui ! Vous le savez, il y a une forme d'exaspération de nos concitoyens à se voir imposer un certain nombre de contraintes,

pousser à la vaccination et responsabiliser toujours davantage celles et ceux de nos concitoyens qui s'y refusent. C'est capital, y compris pour contrer l'exaspération légitime de ceux- ils sont immensément nombreux -qui font l'effort de se conformer aux règles de la vie civique.

Cher président, il faut que nous reprenions la marche des choses. Ce texte est un outil majeur- ce n'est pas le seul -pour lutter contre cette pandémie qui galope. Je le dis au Sénat

Un consensus- non pas global et certes assorti de nuances -s'est dégagé. Nous devons le capitaliser, parce que l'orientation est bonne. Ne confondez pas : le fond est capital. J'ai besoin, la France a besoin de ce texte pour faire progresser la vaccination quelques secondes.

Malheureusement, depuis quelques heures, l'exposé des motifs a changé. Dans l'exposé des motifs tel que je l'ai relu, il est question de protéger la population est pas employé un autre verbe, qui consiste à montrer du doigt, à stigmatiser une partie de la population française. Il est vrai que le

C'est une solidarité, c'est un problème moral, c'est un devoir que l'on peut s'assigner à soi-même vis-à-vis des autres, mais il n'y a pas de règle qui imposerait que l'on soit vacciné.

monsieur le Premier ministre,

Être citoyen, c'est aussi avoir des devoirs. Et de le leur rappeler, c'est tout ce que nous faisons. Nous continuerons, cher président, à faire progresser la vaccination, à « aller vers

La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly, pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste. Monsieur le secrétaire d'État, le peuple mérite autre chose que des insultes, des menaces de mise au ban de la citoyenneté ou des incitations à la fracturation, au clivage, à la haine. Ce peuple, que le président Macron méprise tant, subit sans cesse des injustices graves. Je vais vous en donner un exemple. Alors que le variant omicron frappe notre pays, vous avez fait le choix de maintenir l'entrée en vigueur, au 1 janvier 2022, du forfait de 19,60 euros aux urgences. Ce droit d'entrée, en pleine pandémie, est un non-sens sanitaire, qui va pénaliser de nombreux citoyens. Aujourd'hui, 9 millions de personnes vivent au-dessous du seuil de pauvreté ; 3,8 millions de personnes sont sans mutuelle. Elles n'ont pas les 20 euros dans leur poche, monsieur le ministre ! La priorité n'est-elle pas de lutter contre les déserts médicaux ? Le coeur du problème est là : l'impossibilité, pour nos concitoyens, d'obtenir un rendez-vous avec un médecin, notamment le soir et le week-end, les amène aux urgences.

sont évidemment réelles ; elles le sont depuis de nombreuses années ; elles ont été amplifiées, évidemment, par la crise du covid. Au-delà des grandes déclarations, il est important, à un moment donné, d'objectiver la situation, afin de prendre les mesures les plus adéquates. C'est ce qu'a fait le ministre Olivier Véran, lorsqu'il a annoncé

Nous avons une préoccupation importante au sujet des services d'urgences pédiatriques. Vous avez vu qu'en Seine-Saint-Denis, notamment, un service d'urgences pédiatriques a dû être suspendu au regard de la situation RH. depuis le début de l'année, nous continuons à soutenir les soignants, grâce notamment au doublement de la majoration des heures supplémentaires du temps de travail et grâce à la mobilisation collective du public, du privé et de l'ambulatoire. Quant au forfait patient urgences, en vigueur

aux problématiques que vous avez soulevées.

qui s'appliquera désormais à tous, y compris aux malades en affection de longue durée. Vous allez créer deux catégories de malades : ceux qui auront les moyens de se soigner et ceux qui ne les auront pas et qui vont renoncer aux soins. Inévitablement, ces retards de prise en charge vont aggraver leurs pathologies. Ces femmes et ces hommes viennent-ils saper la solidité du système de santé ? Sont-ils des irresponsables ? Ne seraient-ils plus des citoyens ? Lorsqu'un pays traverse une crise comme celle que nous connaissons, il est du devoir des responsables politiques de garantir l'unité et la cohésion de la Nation, en respectant les citoyens et leur représentant élus. Ce n'est pas la voie que votre président a choisie. La parole est à M. Julien Bargeton, pour le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants. vous adresser mes meilleurs voeux, ainsi qu'à l'ensemble de notre assemblée, aux collaborateurs, aux administrateurs, aux huissiers, à tous les personnels du Sénat qui sont là pour nous et, bien sûr, au Gouvernement, à qui je souhaite une excellente année 2022.

Pour pérenniser ces résultats, il faut investir dans l'avenir et c'est ce que nous faisons. L'avenir, ce sont d'abord les jeunes. En réformant l'apprentissage et en y investissant massivement, nous avons révolutionné l'entrée dans le monde du travail. Avec le contrat d'engagement jeune, nous disons à chacun qu'il peut être accompagné pour trouver sa place sur le marché du travail. L'avenir, c'est aussi la formation de tous. Avec le succès incontestable de Mon compte formation, nous disons aux Français : osez ! C'est ainsi que nous lèverons l'un des verrous du marché du travail dans notre pays, celui de l'adaptation des compétences et des reconversions professionnelles. L'avenir, c'est également de dire aux demandeurs d'emploi de longue durée que le chômage n'est pas une fatalité. C'est pourquoi nous avons doté le plan de réduction des tensions de recrutement de 1,4 milliard d'euros, en plus des 15 milliards d'euros du plan d'investissement dans les compétences. Au-delà, nous voulons valoriser le travail. Il émancipe et il permet de trouver sa place dans la société.

et Républicain. Permettez-moi de présenter à chacun et aux membres du Gouvernement tous nos voeux pour cette nouvelle année. Monsieur le Premier ministre, oui, plaçons-nous au fond du sujet. Votre gestion de la vague actuelle est un échec, car vous avez trop laissé circuler le virus- et je dois dire que c'est très réussi. Depuis six mois, nous avons porté deux propositions fondamentales pour réduire la circulation du virus. Premièrement, la vaccination de toutes et tous, posée comme un principe simple, clair et solidaire : celui de l'obligation vaccinale universelle. C'est un devoir envers les autres, c'est un devoir envers les soignants, qui sont de nouveau submergés, entre désespoir et colère. Avoir refusé une position de principe forte et courageuse pour que le chef de l'État se livre maintenant à une surenchère verbale provocatrice signe un échec. Deuxièmement, la nécessité de réduire fortement la circulation du virus chez les enfants, dans les écoles. Or vous avez choisi, depuis l'automne, de laisser circuler le virus, avec des protocoles improbables, qui déstabilisent les écoles. Nous n'oublions pas que, alors que les cas flambaient au mois de novembre, votre ministre de l'éducation a même osé alléger le protocole. Monsieur le Premier ministre, nous vous proposons d'adopter une stratégie plus respectueuse des Français. Allez-vous instituer, sans vous déguiser et comme le défend maintenant votre prédécesseur, l'obligation vaccinale universelle et alors accepter de débattre, dans l'apaisement, dans le respect du Parlement, des moyens de contrôle et, parmi ces moyens- pourquoi pas ? -d'un passe vaccinal, dont nous sommes prêts à débattre des modalités ? Allez-vous cesser de mener dans les écoles une politique inefficace et qui désempare les parents ?

Et pourtant, il y avait 30 % de personnes hospitalisées en plus. Et pourtant, il y avait un couvre-feu dans le pays ; les restaurants, les bars, les théâtres et les cinémas étaient fermés. C'est grâce à cette couverture vaccinale très large que nous pouvons aujourd'hui tenir dans ces conditions. C'est grâce au passe sanitaire et, demain, au passe vaccinal, que nous atteignons cette couverture très large.

L'une des conséquences visibles de cette situation est la multiplication des vignes en friche, abandonnées par leurs exploitants, qui ne parviennent plus à tirer un revenu décent de la culture de leurs parcelles. Chacune d'entre elles constitue un foyer potentiel pour la prolifération de maladies et de ravageurs de la vigne, comme la cicadelle, porteuse de la flavescence dorée. Pour éviter le dépérissement du vignoble, il est parfois indispensable de traiter ou, si la maladie est déjà présente, d'arracher ces vignes. Mais, alors que traitement et arrachage sont obligatoires dans certains cas point de vue réglementaire, il n'existe aucun moyen de contraindre ou de sanctionner un propriétaire qui ne prendrait pas les mesures rendues nécessaires par la situation sanitaire de ses parcelles. Les syndicats viticoles des vignobles touchés sont inquiets, car les chiffres sont en hausse pratiquement partout. C'est le cas dans le Bordelais, où les services de l'État, en partenariat avec la fédération des grands vins, l'interprofession et les acteurs locaux de la vigne et du vin, ont commencé à constituer sur un territoire de préfiguration, le Blayais, un diagnostic chiffré pour mesurer l'ampleur de la tâche. À l'heure où le recensement agricole montre la diminution constante du nombre de viticulteurs en France, pointant le risque de voir nos paysages viticoles se désagréger, il est indispensable de donner à nos vignerons les moyens de continuer à exercer leur métier, mais aussi de sanctionner les manquements, lorsqu'ils sont avérés. Cependant, l'État lui-même est aujourd'hui dans l'incapacité de savoir à qui appartiennent certaines de ces parcelles à l'abandon, vecteurs de problématiques pour les pour les voisins, d'autant plus s'il s'agit de pépinières viticoles, comme pour les communes. Monsieur le ministre, que prévoyez-vous de mettre en place pour accompagner les viticulteurs français, préserver l'état sanitaire du vignoble et, plus globalement, assurer la survie

votre question me permet de rappeler notre engagement commun au service du secteur vitivinicole, qui est une partie de notre patrimoine culturel, territorial et gastronomique et qu'il nous faut absolument accompagner. Vous m'interrogez sur la multiplication de ce qu'on appelle les vignes laissées en friche. C'est un sujet important de préoccupation partout sur notre territoire,

Territoires. Monsieur le Premier ministre, je vous adresse tout d'abord mes meilleurs voeux, des voeux de concorde, car plus que jamais il faut rassembler les hommes et les femmes de ce monde pour faire face à la pandémie et, au-delà, au dérèglement climatique. Nous sommes fatigués par deux années de pandémie : le système de santé est exsangue ; la société est fracturée comme rarement dans notre histoire ; la situation, en Guadeloupe notamment, est des plus tendues ; la situation économique et sociale est précaire et explosive. La bête immonde se nourrit de la peur, de la colère et de la frustration. Dans ce contexte, votre responsabilité et celle du Président de la République sont plus grandes que jamais. Pourtant, les propos parus dans laissent voir un homme qui ne parvient plus à exercer sa fonction et qui trépigne d'impatience d'en découdre dans l'arène électorale. Il s'égare dans la division avec des propos puérils, indignes de sa fonction. L'heure n'est pourtant pas à la joute, d'autant moins que vous avez choisi de conserver, malgré la campagne présidentielle, la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Monsieur le Premier ministre, merci de rassurer la représentation nationale et de nous préciser en quoi votre stratégie sanitaire ne consiste pas uniquement à « emmerder les non-vaccinés

Vous atteignez les limites de la contrainte et vous n'êtes pas capable de convaincre et d'aller vers les publics les plus éloignés du vaccin. La Seine-Saint-Denis, les quartiers nord de Marseille, les outre-mer ne sont pas des repères d'irresponsables auxquels il faut ôter le statut irrécusable de citoyen. Ce sont les territoires les plus pauvres de la République et leur retard de vaccination est votre échec ! Pour en finir avec la pandémie, le sujet n'est pas uniquement la vaccination de 4 millions de Français ; il s'agit surtout de vacciner encore 4 milliards d'êtres humains ! Soyez à la hauteur de ce moment historique et profitez de la présidence française du Conseil de l'Union européenne

âgées dépendantes (Ehpad) ; elle a été reçue avec satisfaction, mais de nombreux professionnels de l'accompagnement souffrent encore d'un manque de reconnaissance. Les foyers occupationnels et les foyers d'hébergement, qui sont gérés par les départements, n'ont reçu aucune information

et d'entretien et les éducateurs spécialisés sont exclus des mesures de revalorisation, alors que, dans les Ehpad, la totalité du personnel bénéficie de la prime mensuelle de 183 euros net. L'aide sociale à l'enfance et les maisons de l'enfance à caractère social ne bénéficient, quant à elles, d'aucune mesure de revalorisation.

très difficiles à justifier auprès des employés et des syndicats. Les salariés sont de plus en plus nombreux à vouloir changer d'établissement pour bénéficier de meilleures conditions de travail. La conférence des métiers et de l'accompagnement social et médico-social, annoncée pour le 15 janvier, a été reportée. Madame la ministre, pour un principe d'équité, tous les employés d'établissements financés par les ARS ou les départements devraient bénéficier d'une revalorisation salariale financée par l'État. Pourriez-vous nous préciser votre feuille de route pour répondre aux demandes d'équité salariale de l'ensemble des personnels des secteurs sociaux et médico-sociaux ?

La mission conduite par M. Laforcade a permis, en février, d'obtenir une première extension pour les structures rattachées aux établissements publics de santé et les Ehpad relevant de la fonction publique hospitalière. Un deuxième accord d'extension est intervenu en octobre pour les soignants des structures publiques non rattachées à un établissement public. Tous les personnels non médicaux des établissements financés par l'assurance maladie bénéficient de cette revalorisation. Au 1 janvier de cette année, 66 000 professionnels du secteur du handicap et de l'accompagnement sont désormais concernés.

La parole est à Mme Christine Lavarde, pour le groupe Les Républicains.

ont pris connaissance du nouveau protocole sanitaire. Mardi matin, c'est en écoutant une interview de Gabriel Attal à la radio que ces mêmes enseignants ont pris connaissance du fait qu'ils auraient l'obligation d'accueillir les enfants des personnels soignants, lorsque les classes seraient fermées. Mais rien n'a été dit à ce jour pour les enfants de moins de

comment expliquer qu'un enfant de 3 ans scolarisé en classe de maternelle revient à l'école s'il est cas contact, à partir du moment où il prouve qu'il a un test négatif, et que ce même enfant, toujours âgé de 3 ans, mais accueilli dans un établissement de petite enfance, doit subir une « quarantaine » de 17 jours ?

peu de bon sens et éclairer les familles sur ce qui va advenir des enfants de moins de 3 ans

et le pragmatisme sont ce qui guide le Gouvernement depuis le début de cette crise sanitaire il y a deux ans. Ce qui nous guide aussi depuis deux ans, c'est le souci d'assurer

: gouverner, c'est prévoir ; ne rien prévoir, c'est courir à sa perte

la taxinomie- ou taxonomie -européenne permet aux différents secteurs économiques d'avoir accès à des taux d'emprunt préférentiels sur les marchés financiers. Cette taxinomie sera donc un levier structurant pour soutenir les investissements importants qui sont nécessaires pour atteindre nos objectifs de réduction d'émission de gaz à effet de serre de 55 % d'ici à 2030 et de neutralité carbone en 2050. Pour l'agriculture française, qui aura un rôle majeur à jouer, les enjeux sont considérables pour financer à des coûts minimisés les investissements qui s'inscrivent dans la stratégie dite « de la ferme à la fourchette », laquelle constitue le volet agricole du Pacte vert pour Monsieur le ministre, alors que la présidence française du Conseil de l'Union européenne s'ouvre, ma question sera triple. Premièrement, quelle est l'ambition politique de la France en matière de finance durable de l'agriculture ? Allez-vous proposer et négocier des critères auprès de la Commission européenne pour que les investissements des agriculteurs français soient éligibles à cette finance durable ? Deuxièmement, si tel est le cas, pouvez-vous nous donner des exemples concrets pour que les agriculteurs qui nous écoutent en soient informés ? Quelles filières y auront accès ? Les services environnementaux auxquels je suis attaché seront-ils, par exemple, concernés ? Troisièmement, le plan stratégique national français, dont nous ne connaissons officiellement pas grand-chose à ce jour, intégrera-t-il ce sujet, qui conditionne en partie la compétitivité durable de l'agriculture française ? Si oui, quel calendrier envisagez-vous ?

Daniel Gremillet, pour le groupe Les Républicains. C'est avec une réelle anxiété que nous avons pris connaissance du projet d'acte délégué sur la taxonomie verte proposé par la Commission européenne, car il est en retrait par rapport à la résolution adoptée par le Sénat le 7 décembre L'énergie nucléaire serait assimilée non pas à une activité durable, mais à une activité transitoire. Elle serait mise sur le même plan que le gaz naturel. C'est une complète aberration en ce qui concerne le climat, car les émissions sont sans commune mesure écologique), une centrale nucléaire émet 6 grammes de CO2 par kilowattheure, contre 418 grammes pour une centrale à gaz. C'est aussi un sérieux revers vis-à-vis de notre partenaire allemand. L'énergie nucléaire serait soumise à une information spécifique, ne garantissant pas la neutralité technologique avec les autres énergies décarbonées. Elle ne serait intégrée que dans un an, alors que la taxonomie est applicable depuis le 1 janvier comment justifier un tel décalage ? Les rénovations de centrales seraient éligibles jusqu'en 2040 et leur construction jusqu'en 2045, alors que tous les scénarios démontrent que les besoins d'investissement vont bien au-delà de 2045. Ce statut transitoire est un non-sens au regard de l'objectif cardinal visé par la taxinomie : l'atteinte de la neutralité carbone. Aussi, madame la ministre, ma question est simple : quelle est la position du Gouvernement sur ce projet ? Que compte-t-il faire pour obtenir un statut, une information, un délai et des conditions plus favorables pour l'énergie nucléaire ?

Mesdames, messieurs les sénateurs, c'est désormais chose faite ! C'est très exactement ce qui vient de se passer, car le texte aujourd'hui proposé par la Commission européenne- il n'est pas encore adopté, je le rappelle -précise très clairement que le nucléaire est une énergie bas-carbone et sûre, ce qui nous donne les outils de financer nos projets dans le cadre de la finance durable. C'est une étape décisive pour la filière nucléaire et ses 220 000 professionnels. C'est une étape décisive pour notre mix énergétique, dans lequel le nucléaire garantit une énergie stable, bon marché et accessible. C'est une étape décisive pour notre indépendance énergétique. On voit bien aujourd'hui, alors que les prix du gaz

font partie de la colonne vertébrale de l'Union européenne. Il dissuadera les financeurs de s'engager dans la filière nucléaire. Comment voulez-vous inciter les chercheurs et les jeunes à s'engager dans une filière transitoire ? transitoire ? Cela pèsera lourdement sur la compétitivité de notre économie et le pouvoir d'achat des ménages. Où est le retour en grâce du nucléaire annoncé à l'automne par le Président de la République ? La présidence française du Conseil de l'Union européenne commence bien mal

Une disposition, cependant, pose problème : elle impose, en niveau 3, qu'en l'absence d'un professeur non remplacé les enfants ne sont plus répartis dans les autres classes ; ils ne sont tout simplement plus accueillis à l'école. Pour reprendre le choix lexical du moment, cette règle « emmerde » tous les parents, vaccinés ou non. Pour chaque absent, vingt-cinq familles apprennent à huit heures vingt qu'elles doivent garder leur enfant ; la vie des familles est précarisée, la continuité pédagogique et sociale rompue. Les parents, assignés à résidence, ne pouvant travailler, l'économie est perturbée, sans que la covid en soit nécessairement la cause.

les mêmes enfants sont mélangés en dehors de l'école, en famille, lors des activités associatives. Ils le sont aussi sur les temps périscolaire, malgré les règles de zonage, d'horaires, malgré les tentatives de maintien en groupes « classe » mis en place par les collectivités. Quoi qu'il en soit, la répartition dans les autres classes est traçable. Bien sûr, le remplacement de chaque professeur absent demeurerait la meilleure solution. Néanmoins, ce n'est pas nouveau, peu d'absents sont remplacés, et toujours avec un temps de latence. Les recrutements que vous avez engagés porteront au mieux le taux de 9 % à 15 % des effectifs. C'est loin de répondre au problème posé immédiatement par le protocole. Je vous sais soucieux de maintenir la continuité pédagogique et l'école ouverte. Alors, monsieur le ministre, quand allez-vous supprimer cette règle de non-accueil à l'école des enfants dont les professeurs absents ne sont pas remplacés ?

directeurs d'école, chefs d'établissements, et tous les personnels, y compris des collectivités locales, que je salue, parce que nous savons tous que c'est dur pour eux, comme c'est dur pour les parents d'élèves. Est-ce que je vais nier que le mois de janvier sera difficile ? Bien sûr que non ! Le mois de janvier est et sera difficile. Les situations que vous décrivez sont bien réelles et très compliquées.

Il est impossible de dire quel sera le pic d'absences, mais il ne devrait pas dépasser normalement 15 %. En tout cas, nous déployons actuellement des moyens pour aller au-delà des 9 % de moyens de remplacement, c'est-à-dire aux alentours de 12 d'absence cette semaine, tel que nous pouvons le constater, est de 7 %, donc nous sommes en ce moment en mesure de remplacer, avec, bien entendu, des exceptions. Il y en a, je le reconnais, mais nous sommes bel et bien en situation de mener cette politique de l'école ouverte, qui correspond au désir de tous,

tous les Français. Ma question s'adresse à M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Sans jamais avoir été une colonie britannique, le Gabon vient d'annoncer, par la voix de son président, son adhésion en 2022 au Commonwealth. Le Gabon se tourne vers un autre monde, à savoir la sphère anglophone. Il n'est pas le seul à se détourner de nous. À l'heure du Brexit, ils sont nombreux à souhaiter s'ouvrir à de nouveaux partenaires, qu'ils jugent plus intéressants et plus flexibles en matière économique, géopolitique et de développement le Cameroun, le Rwanda, le Gabon, que j'ai cité, le Togo et, peut-être demain, le Maroc, qui se sentirait, selon un ancien ambassadeur marocain, « étriqué » dans la francophonie. Monsieur le ministre, l'Hexagone perd du terrain, notamment au profit de l'influence britannique à travers l'organisation du Commonwealth et des accords commerciaux de libre-échange plus avantageux. Un autre phénomène, bien plus inquiétant encore, témoigne de l'affaiblissement de la France : il s'agit, bien sûr, de l'irruption de la société militaire privée russe Wagner au Mali, comme dans beaucoup d'autres pays en crise. Comment expliquer que les autorités de transition à Bamako lui accordent aujourd'hui davantage leur confiance pour assurer leur sécurité qu'à la France, qu'elle avait pourtant appelée à son secours voilà dix ans ? Comment expliquer que Wagner arrive à faire oublier ses échecs cuisants et ses exactions dans d'autres États africains, pendant que se répand un sentiment anti-français de plus en plus fort dans la zone sahélienne ? Des décennies d'interventions sous mandats juridiques internationaux et des décennies d'aide au développement pour maintenir la paix et éviter des affrontements communautaires sanglants sont aujourd'hui balayées par une diplomatie d'observation. J'en viens à ma question : monsieur le ministre, quelle est la stratégie du Gouvernement pour réinvestir le « champ informationnel », que vous avez vraisemblablement délaissé, voire oublié ? La La parole est à M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Monsieur le sénateur Cédric Perrin, je ne partage pas votre point de vue. Depuis plusieurs mois, les seules initiatives majeures qui ont été prises à l'égard de tout le continent africain, avec les Africains, viennent de la France. Je vais vous le démontrer, mais vous le savez bien, puisque j'en parle régulièrement avec vous à la commission des affaires étrangères du Sénat. D'abord, le 18 mai dernier, le Président de la République a réuni à Paris une très grande partie des chefs d'État africains, anglophones, francophones ou lusophones, pour aborder avec eux le plan de relance économique pour l'Afrique et permettre la mobilisation de 100 milliards de dollars de droits de tirage spéciaux en faveur de l'Afrique. Jamais cela n'aurait été possible sans la France.

et combattent avec nous contre l'arrivée de Wagner en Afrique occidentale. C'est aussi pour cette raison que nous allons engager ce avec l'Afrique, sous la présidence française de l'Union européenne, les 17 et 18 février prochains à Bruxelles. réunir les ministres des affaires étrangères de l'Union européenne, en présence de M. Moussa Faki, le président de la Commission de l'Union africaine, la semaine prochaine. La France est respectée, la France est reconnue, la France est attendue en Afrique La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ils parleront de notre sécurité, sans que nous soyons présents ... Depuis plusieurs semaines, nous assistons à une montée des tensions et à une augmentation des mouvements aux frontières de l'Ukraine, dont la Russie a déjà violé l'intégrité territoriale. Depuis de nombreux mois, Moscou a bloqué les initiatives du format « Normandie », lancé sur l'initiative de la France et de l'Allemagne en juin 2014 pour trouver une issue à la guerre à l'est de l'Ukraine. Ce format ne mobilisait que des Européens. Aujourd'hui, le président de la Fédération de Russie pose des conditions nouvelles censées être indispensables à la sécurité de son pays. Il pose des conditions qui portent atteinte au droit de chaque État européen de définir par lui-même sa politique étrangère et sa politique de sécurité. Il pose des conditions qui violent le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Il pose des conditions à un moment où les évolutions constatées à l'intérieur de son pays inquiètent de nombreux observateurs. Dans quelques jours, Moscou et Washington parleront de nous sans nous. Nous voilà donc revenus à l'avant-1989, à cette Europe de Yalta, cette Europe divisée, cette Europe mise sous tutelle, que nous ne voulons pas revoir. Pendant des années, du président Charles de Gaulle au président François Mitterrand, notre politique étrangère n'a eu de cesse de vouloir sortir l'Europe de ses fractures et de ses dépendances, de rendre à chaque peuple européen sa liberté. En 1989, les peuples européens ont gagné le droit de dire : « Rien sur nous sans nous ! » Ce droit constitue le fondement de notre indépendance stratégique. Nous ne pourrons rien construire en Europe si un seul pays ne dispose pas de sa totale liberté. Nous ne pourrons rien construire si ce droit est violé. Monsieur le ministre, alors que commence la présidence française du Conseil de l'Union européenne, comment envisagez-vous de défendre cette autonomie stratégique,

Préalablement à ces rencontres, la Russie a déposé sur la table sa conception des paramètres de la sécurité européenne. Face à cela, nous devons avoir, à mon sens, trois réactions. Premièrement, nous ne devons pas refuser la discussion avec la Russie. Ce dialogue peut contribuer à renforcer notre sécurité, mais il doit se faire sur la base de paramètres que nous jugeons pour nous pertinents et qui sont conformes à nos intérêts collectifs de sécurité. Or plusieurs des propositions russes ne sont pas compatibles avec les principes fondamentaux de la sécurité et de la stabilité européennes, auxquels vous faisiez allusion, et qui étaient ceux de l'accord

la sécurité européenne ne saurait se discuter sans leur pleine implication. Tel sera d'ailleurs le sujet des premières réunions des ministres des affaires étrangères et des ministres de la défense, qui vont se tenir conjointement à Brest la semaine prochaine, dans le cadre de cette séquence, pour affirmer notre position. Enfin, troisièmement, le dialogue avec la Russie ne doit pas nous faire oublier la fermeté nécessaire que nous devons manifester sur la crise ukrainienne : nécessité de la discussion en format « Normandie », ce que chacun reconnaît, sauf la Russie aujourd'hui- les États-Unis sont bien sur cette position ; mise en oeuvre des accords de Minsk ; menace de conséquences massives s'il y avait une nouvelle atteinte à l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Telle est notre position. Elle est claire et elle va être répétée au sein de toutes les instances internationales dans les jours qui viennent. La parole est à Mme Catherine Dumas, pour le groupe Les Républicains. de l'Europe et des affaires étrangères, la réforme voulue par le Président de la République et visant à supprimer les grands corps de l'État au profit d'un corps unique d'administrateurs de l'État vient de connaître son premier développement avec la création de l'Institut national du service public. Cette réforme va s'appliquer au ministère de l'Europe et des affaires étrangères, et elle inquiète légitimement nos diplomates : 800 d'entre eux sont concernés par la disparition progressive des corps de conseiller des affaires étrangères et de ministre plénipotentiaire à partir de 2023. Aujourd'hui issus de l'ENA, voire du prestigieux et sélectif concours d'Orient, ces serviteurs de l'État embrassent cette carrière par vocation, pour servir la France à l'étranger. l'étranger. Le métier de diplomate n'est pas celui de préfet ou d'inspecteur général des finances : être diplomate, c'est posséder des compétences de négociation, une expérience sur le terrain acquise au fil des années et des postes. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous confirmer le maintien du concours du cadre d'Orient, qui fait la réputation du plus vieux service diplomatique au monde, et nous préciser si les ambassadeurs seront toujours nommés sur votre proposition ?

j'ai veillé à pouvoir articuler les priorités de la réforme de la haute fonction publique, souhaitée par le Président de la République, avec ces nécessités. J'ai obtenu sur ces orientations le soutien plein et entier du Premier ministre. Madame la sénatrice, je peux le concours d'Orient, qui restera une voie d'accès directe et spécifique au Quai d'Orsay, sera maintenu. Le ministère en maîtrisera les modalités d'organisation et les lauréats continueront à être recrutés en raison de leur profil spécialisé, s'insérant dans une filière professionnelle clairement identifiée. la revalorisation des parcours et des carrières des agents qui ont rejoint le ministère comme secrétaire des affaires étrangères sera renforcée. En outre, le Premier ministre a bien voulu garantir que les conseillers des affaires étrangères ou ministres plénipotentiaires

comme cela se produit dans certains pays. Des postes diplomatiques prestigieux risqueraient d'être occupés par des non-diplomates, ce qui, bien entendu, n'est pas souhaitable. Nous possédons le deuxième réseau diplomatique au monde, un monde aujourd'hui en plein vertige, les crises internationales se multipliant. Il n'est vraiment pas opportun d'affaiblir la France dans de telles circonstances. La parole est à M. Jean-Michel Arnaud, pour le groupe Union Centriste.

Pour l'électricité, alors que le mégawattheure coûtait 69 euros au printemps dernier, il a atteint 168 euros le 5 octobre dernier, et plus encore dans les mois qui ont suivi. Face à la volatilité des prix, le Gouvernement a mis en place un bouclier tarifaire à destination des particuliers : le fameux chèque inflation de 100 euros. En revanche, aucune mesure n'a été prise pour soutenir les communes et les intercommunalités. Si ces dernières ont jusqu'alors été préservées par ces mouvements de marché grâce à des contrats pluriannuels à prix fixes, nombre d'entre elles renouvellent actuellement les contrats avec les fournisseurs d'électricité et ont pu constater l'envolée des coûts.

Cette situation est d'une gravité exceptionnelle pour les finances des collectivités territoriales et la qualité des services dus à nos populations. Les citoyens et contribuables subissent un double préjudice : des fermetures forcées d'équipements publics et des hausses de prélèvements obligatoires lorsque les fermetures administratives sont impossibles, pour des raisons d'hygiène publique par exemple. Je pense aux stations d'épuration ou de traitement des eaux. Ma question est la suivante : face à l'augmentation non maîtrisable du coût de l'énergie

Le principal outil de protection des consommateurs- je reviendrai évidemment sur les collectivités -, c'est une baisse temporaire de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TICFE) à partir du 1 février 2022,

Nous allons en tout cas veiller à ce que les collectivités puissent vraiment bénéficier de cette baisse temporaire de la TICFE, de manière à amortir une partie de l'augmentation des prix de l'énergie. Votre question me permet aussi de souligner combien il a été utile, pendant toute cette période de crise que nous traversons, de préserver les ressources des collectivités. C'est ce qui avait guidé nos choix lorsque nous avons mis en place un filet de protection en matière de recettes fiscales et domaniales en 2020, et en matière de recettes fiscales en 2021. De la même manière, c'est ce qui a guidé nos choix lorsque nous avons mis en place

sur la baisse de l'épargne brute, ce qui permettra aussi d'apporter des réponses à des régies fortement concernées par l'augmentation de l'électricité. Nous restons évidemment très vigilants. Les collectivités, comme l'ensemble des acteurs- particuliers, industriels, acteurs économiques connaissent des difficultés liées à l'augmentation du prix de l'énergie et nous mettons en oeuvre des mesures, que je viens de détailler, pour un coût qui pourra représenter entre 12 milliards et 15 milliards d'euros par an. Vous admettrez avec moi que c'est considérable. La parole est à M. Jean-Michel Arnaud, de réponse, monsieur le ministre. Cela étant, la notion de bouclier tarifaire mériterait d'être précisée, parce que, dans la pratique, les collectivités qui sont en train de négocier, en particulier avec l'opérateur historique EDF,

La séance est reprise. J'informe le Sénat qu'une candidature pour siéger au sein de la délégation sénatoriale à la prospective a été publiée. Cette candidature sera ratifiée si la présidence n'a pas reçu d'opposition dans le délai d'une heure prévu par notre règlement. J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d'examiner les dispositions restant en discussion du projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d'exercice de cette représentation et portant habilitation du Gouvernement à compléter par ordonnance les règles organisant le dialogue social avec les plateformes est parvenue à l'adoption d'un texte commun.

Mes chers collègues, je vous rappelle que le port du masque est obligatoire dans l'hémicycle, y compris pour les orateurs s'exprimant à la tribune, conformément à la décision adoptée par la conférence des présidents le 1 décembre dernier. J'invite par ailleurs chacune et chacun à veiller au respect des gestes barrières. Dans la discussion générale, la parole est à M. Christian Cambon,

collègues, avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à remercier le président du groupe Les Républicains, M. Bruno Retailleau, d'avoir permis l'inscription rapide de ce projet de résolution à l'ordre du jour de notre assemblée.

D'une part, le Sénat trouve ainsi aujourd'hui une nouvelle occasion de montrer son engagement pour la paix et pour la résolution de ce que l'on appelle souvent les « conflits gelés », ces dossiers si complexes et douloureux qu'ils ont fini par sembler inextricables. D'autre part, si nous avons une ambition indo-pacifique, c'est bien au travers de sujets concrets comme celui-ci que nous devons donner l'image d'une France pleinement actrice des dossiers de cette région du monde.

L'Union soviétique boycottait alors le Conseil de sécurité des Nations unies, en raison de la non-reconnaissance de la République populaire de Chine par celles-ci, Taïwan occupant alors le siège chinois au Conseil. C'est ce qui a permis l'adoption sans opposition

C'est ainsi qu'a été autorisée l'intervention militaire en Corée, qui s'est déroulée de juin 1950 à juillet 1953. La France y a pris toute sa part, membre fondateur de l'ONU et membre permanent du Conseil de sécurité. Elle a immédiatement envoyé un bâtiment de guerre prélevé sur nos forces maritimes d'Extrême-Orient, l'aviso, distingué en 1952 d'une citation présidentielle de la République de Corée. Notre pays a également pourvu à la formation d'un contingent de forces terrestres : le bataillon français de l'ONU, constitué de 1 017 volontaires venus tant de régiments d'active que des réserves, et placé sous le commandement du fameux lieutenant-colonel Monclar.

Il a reçu deux citations présidentielles de la République de Corée, trois citations présidentielles des États-Unis, et a été cité cinq fois à l'ordre de l'armée française. Nous pouvons aujourd'hui rendre hommage

Une alliance militaire a été signée entre les États-Unis et la Corée du Sud en 1953, aux termes de laquelle 29 000 soldats des forces armées des États-Unis demeurent stationnés en Corée du Sud ; des exercices militaires bilatéraux se tiennent régulièrement afin de faire face à une éventuelle attaque nord-coréenne. Cette situation, qui dure depuis près de soixante-dix ans, constitue de fait un obstacle à la négociation d'un traité de paix. Il y a donc lieu de promouvoir

À cette fin, la présente proposition de résolution invite le Gouvernement à prendre les initiatives diplomatiques nécessaires dans cette perspective.

Les tentatives de reprise des discussions entre les deux Corées sont régulièrement interrompues par les velléités de Pyongyang de se doter de l'arme nucléaire, voire d'un arsenal balistique de longue portée dont il tente de démontrer la réalité au travers d'essais volontairement spectaculaires. La Corée du Nord fait valoir ses positions ; alors, affirmons les nôtres, en faveur de la fin de la guerre et de la dénucléarisation de la péninsule coréenne deuxième point où la parole de la France est attendue par nos amis coréens. La dénucléarisation de la péninsule ne sera sans doute pas possible tant que la fin de la guerre ne sera pas déclarée. Nous sommes tous d'accord sur le fait que cette dénucléarisation doit être la plus large, la plus vérifiable et la plus sûre possible. C'est l'un des buts de cette proposition de résolution, telle que nous l'avons rédigée en lien avec nos collègues et amis coréens. Ce texte vient donc appuyer les objectifs des résolutions des Nations unies.

Alors que le régime de la Corée du Nord tente régulièrement d'isoler les initiatives de la Corée du Sud, il est essentiel que nous affirmions notre solidarité et notre soutien sans faille et indéfectible à la démocratie coréenne.

À l'heure où la France comme l'Union européenne entendent mettre en oeuvre une politique indo-pacifique, il est essentiel que nous le traduisions par des actes. Nos positions diplomatiques ne peuvent se limiter à l'affirmation d'ambition sans traduction concrète. Une diplomatie, ce sont des paroles, mais ce sont aussi des actes. Monsieur le ministre, je sais que nous nous rejoindrons sur ce point.

Il paraît donc peu probable que la France soit partie à la signature d'une déclaration de fin de la guerre. En revanche, il est ici proposé que nous agissions pour la reconnaissance par la communauté internationale, et notamment par les Nations unies, de cette déclaration de fin de guerre. De même, la France, qui dialogue avec tous- c'est une de nos grandes forces -, est invitée à engager une conversation avec les parties susceptibles de signer cette déclaration de fin de guerre : Corée du Nord, Corée du Sud, États-Unis et Chine. Nous avons là un rôle à tenir en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies et en tant que nation de l'Indo-Pacifique. Monsieur le ministre, mes chers collègues, voilà donc l'objet de cette proposition de résolution. Je pense que son adoption adressera un signal fort d'intérêt pour la Corée du Sud et de soutien à cette nation. Elle traduira aussi le caractère concret de notre engagement dans la zone indo-pacifique. S'impliquer dans cette zone, ce n'est pas seulement défendre les intérêts directs de notre pays, ses territoires ou ses eaux : c'est aussi renouveler l'engagement de la France pour le droit international, pour le respect des frontières, pour le respect du droit de la mer et, finalement, pour la paix. Oui, même lorsque la situation paraît figée, la paix mérite que l'on remette inlassablement l'ouvrage sur le métier, pour tenter d'avancer. C'est tout l'esprit de la proposition de résolution que j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je suis très heureuse, en tant que présidente du groupe d'amitié France-Corée du Sud, que notre assemblée examine aujourd'hui cette proposition de résolution appelant le Gouvernement à oeuvrer à l'adoption d'une déclaration de la fin de la guerre de Corée.

qui a en tête que les combats ne sont que provisoirement suspendus et que la péninsule coréenne est officiellement toujours en état de guerre ? La convention d'armistice signée de façon temporaire le 27 juillet 1953

plus de 800 000 morts parmi les militaires coréens, nordistes et sudistes confondus, des dizaines de milliers parmi les forces de l'ONU qui sont alors intervenues,

donc omniprésents ; notre groupe d'amitié l'a très fortement ressentie, presque physiquement, lorsque nous nous sommes rendus en Corée du Sud au mois de septembre dernier, à l'invitation de l'Assemblée nationale de de Corée. Vivette Lopez, Olivier Jacquin, Catherine Procaccia et moi-même, qui présidais la délégation, avons en effet été frappés par la sensibilité du sujet en Corée que nous avons tendance à voir la situation actuelle comme un produit de l'histoire qui se serait figé avec le temps, cette situation reste vécue par la population et les dirigeants sud-coréens comme un enjeu existentiel. Je veux dire par là que les Coréens du Sud ont le sentiment que leur avenir, leur existence future en dépendent. visite de la DMZ, la zone démilitarisée séparant les deux Corées, qui constitue en réalité l'un des endroits où le degré de tension entre deux États est le plus élevé sur la planète, a permis à notre délégation d'éprouver pleinement cette dimension si prégnante dans la société coréenne d'aujourd'hui. L'état de guerre qui perdure et la coexistence avec leur voisin nord-coréen

témoignage de ces hauts faits d'armes, nous avons visité le cimetière du mémorial des Nations unies en Corée, situé à Busan, la deuxième ville du pays. Au cours d'une cérémonie extrêmement émouvante, notre délégation a déposé une gerbe dans le carré français du cimetière, qui compte 46 tombes individuelles. Cet appui de la France à l'armée sud-coréenne nous a été constamment rappelé lors de nos rencontres officielles, nos amis sud-coréens l'ayant sans doute beaucoup plus à l'esprit que nous-mêmes. Ce fut le cas lors de notre rencontre avec mon homologue, le président du groupe d'amitié interparlementaire Corée-France, M. Jung Sung-ho, et des membres de ce groupe. Cet attachement historique à la France nous donne une légitimité particulière pour intervenir dans ce dossier, et ce d'autant plus que d'autres éléments plus contemporains s'y ajoutent, comme il a été rappelé par M. Cambon. Ce contexte étant posé, la proposition de résolution que nous examinons aujourd'hui me semble aller dans le bon sens, qui est aussi le sens de l'histoire celui de la conversion d'une convention d'armistice précaire et réversible en un état de paix durable à travers la conclusion d'un véritable traité de paix entre les belligérants. En se prononçant pour une déclaration officielle de la fin de la guerre de Corée, notre assemblée enverra un signal politique à un moment où celui-ci est plus que jamais nécessaire, du fait du nouveau refroidissement des relations entre les deux Corées, mais aussi entre la Corée du Nord et les États-Unis, qui jouent bien sûr un rôle central dans ce dossier. À l'heure où le dialogue entre les principaux acteurs du conflit stagne, il paraît utile de rappeler l'horizon vers lequel les efforts et la concertation doivent porter, à savoir le rétablissement d'une paix durable sur l'ensemble de la péninsule coréenne. Cet objectif a d'ailleurs été plusieurs fois proclamé par les deux belligérants principaux, lors des sommets intercoréens de 2000, 2007 et 2018.

S'il nous faut donc oeuvrer en faveur de la reconnaissance de la fin de la guerre de Corée, encore faut-il que ce processus respecte certaines conditions, que je crois bon de rappeler ici. Tout d'abord, notre pays, qui a pris part au conflit et qui est présent auprès du commandement des Nations unies, devra, même s'il n'a pas été signataire de la convention d'armistice, être associé d'une façon ou d'une autre aux futures négociations du traité de paix. Ensuite, il importe de veiller au maintien en place du commandement des Nations unies, doté d'un nouveau commandant depuis cet été. Cette structure a en effet joué un rôle majeur, sous mandat de l'ONU, pour mettre en oeuvre l'accord d'armistice et veiller aux conditions du maintien de la paix entre les deux Corées. Enfin et surtout, l'objectif de dénucléarisation que mentionne la proposition de résolution devra être aligné sur les objectifs onusiens en la matière, propres à garantir un démantèlement complet, vérifiable et irréversible des programmes nord-coréens. Pour conclure, sous réserve de ces quelques conditions d'interprétation du texte qui nous est soumis aujourd'hui, je voterai donc en faveur de son adoption. Il est en effet temps, pour reprendre les propos attribués à Cicéron, que les armes le cèdent à la toge et que les Coréens, du Sud comme du Nord, puissent vivre sur la même péninsule dans une paix

le sujet qui nous occupe aujourd'hui ne doit pas nous laisser indifférents. En effet, c'est sur ce continent où les poids lourds démographiques et économiques se côtoient que la paix devra être protégée avec le plus de détermination dans les années qui viennent. de soixante-dix ans après la fin des opérations militaires sur la péninsule coréenne, ce conflit est loin d'être gelé sur le tracé du 38 parallèle : les programmes d'armement nord-coréens se poursuivent, comme le rappelle le lancement par Pyongyang d'un premier missile supposément hypersonique, le 19 octobre dernier.

Souvenons-nous également de la crise de 2018 : à la suite de l'essai nucléaire de Pyongyang et du lancement d'un missile de longue portée, Donald Trump, alors président des États-Unis, avait envisagé des frappes préventives sur la Corée du Nord pour faire cesser son programme nucléaire.

historique par la Corée du Sud. Nous sommes loin de cet optimisme aujourd'hui ! Depuis le sommet de Hanoï, en 2019, où les talents de diplomate de Donald Trump n'ont permis aucune avancée dans les négociations, le dialogue est en suspens et avec lui les espoirs d'apaisement. Tristes voeux de Nouvel An que ceux de Kim Jong-un, qui déclarait le 1 janvier vouloir encore renforcer ses capacités de défense nationale ! Je suis donc convaincu qu'il serait irresponsable de ne pas nous mobiliser pour encourager toutes les parties à la guerre de Corée à s'accorder enfin sur une déclaration de paix. Nous voterons donc bien évidemment en faveur de cette proposition de résolution. Cette position est par ailleurs motivée par l'inquiétude qui est la nôtre face à la militarisation actuelle de la zone indo-pacifique et aux stratégies croissantes de contestation de la Chine dans cette zone, qui sont partie intégrante du problème coréen. Retrouver le chemin de la table des négociations ne se fera bien sûr pas d'un claquement de doigts. Si nous entendons les dirigeants nord-coréens affirmer leur ouverture à la reprise du dialogue, nous savons que les demandes qu'ils adressent aux États-Unis comme condition de cette reprise sont irréalistes, car la question nucléaire reste le sujet de dissensions majeures. Le programme de développement des capacités nucléaires nord-coréennes, qui semblait ralenti depuis le dialogue de 2018, a été l'un des points d'achoppement ayant mené à l'échec des négociations de 2019 ; l'arrêt temporaire d'un complexe nucléaire produisant du plutonium, qui constituait une première avancée, semble désormais appartenir au passé si l'on en croit les alertes émises par l'Agence internationale de l'énergie atomique au mois d'août dernier. La reprise de ces activités d'enrichissement nucléaire à destination militaire constitue une violation flagrante des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU elle menace toute la région, notamment le Japon, dont il convient de rappeler qu'il est l'un de nos principaux partenaires stratégiques en Asie et dans l'Indo-Pacifique. Nous devons donc continuer à porter avec détermination notre souhait de voir les parties à la guerre de Corée se retrouver autour de la table des négociations tout particulièrement le faire auprès des pays amis que sont la Corée du Sud et les États-Unis. Nos amis états-uniens doivent faire face à leurs responsabilités et démontrer une vraie volonté politique d'arriver à une déclaration de paix, qui pourrait constituer un signal encourageant pour l'arrêt du programme nucléaire de la Corée du Nord. Ce début d'année 2022 est une occasion inespérée de voir se réaliser ce souhait, alors que le président sud-coréen Moon Jae-in, très attaché au rapprochement avec la Corée du Nord, arrive à la fin de son mandat et que le régime nord-coréen fait face sans vaccin à une pandémie non maîtrisée, mais aussi à une récession sans précédent accompagnée d'une énième crise alimentaire. En cette année qui verra la première conférence du traité sur l'interdiction des armes nucléaires (TIAN) et la dixième conférence du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), il est nécessaire d'oeuvrer à la résolution de ce dernier vestige de la Guerre froide pour donner davantage de force au mouvement mondial pour le désarmement nucléaire. C'est donc tout naturellement que les écologistes invitent le Gouvernement français à agir en ce sens. Très

Il est en effet plus que jamais nécessaire d'abaisser le niveau persistant des tensions entre les deux Corées, ainsi qu'entre la Corée du Nord et les États-Unis, dans une région indo-pacifique elle-même sous tension, et d'ouvrir enfin la voie à un traité de paix définitif pour toute la péninsule coréenne.

de demander aux autorités de notre pays de prendre des initiatives politiques en vue d'instaurer une paix durable entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, assorties de mesures de réduction des arsenaux nucléaires. Tout nous y invite la situation dans la région et la tension nouvelle dans le monde, alors que l'escalade militaire et nucléaire est repartie de plus belle. Entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, nous le savons, la paix n'a jamais été scellée. Depuis près de soixante-dix ans, la péninsule coréenne est coupée en deux, son peuple écartelé. Dix millions de familles restent séparées par la frontière. Les plaies d'un conflit qui a fait cinq millions de morts et de blessés et six millions et demi de réfugiés ne sont pas refermées. Un traité de paix marquerait un pas historique. Depuis 2017, les discussions ont repris, mais les dirigeants nord et sud-coréens successifs et les dirigeants états-uniens ont soufflé tour à tour le chaud et le froid, laissant un temps espérer l'avancée du dialogue, envoyant à d'autres moments des signaux d'alerte et d'escalade. Nous assistons alternativement à des réchauffements et à des coups d'arrêt. Au total, la région reste une inquiétante poudrière. Est-il possible de progresser réellement vers une paix durable ? Oui,

L'échéance olympique de 2018 à Pyongyang avait permis des échanges de lettres et- image symbolique ! -la création d'une équipe commune de hockey sur glace. Le sommet intercoréen et la déclaration de Panmunjom, soutenue quelques mois plus tard par la déclaration coréo-états-unienne de Singapour, ont ouvert des perspectives. Enfin, la réouverture des canaux diplomatiques entre le nord et le sud au mois de juillet dernier mérite d'être soulignée. Toutefois, malgré ces marqueurs forts, les zones d'ombre restent elles aussi majeures. Le sommet de Hanoï en 2019 entre Donald Trump et Kim Jong-un a montré que la tension demeurait forte entre Pyongyang et Washington. Les États-Unis veulent plus que le seul démantèlement du complexe de Yongbyon. Pyongyang ne peut accepter le renvoi à des discussions ultérieures de la suspension des sanctions internationales. Surtout, la reprise de la course aux armements, au sud comme au nord,

partie du cercle très fermé des pays disposant d'avions de chasse supersoniques. La Corée du Nord n'est pas en reste. Pyongyang souhaite développer son arsenal nucléaire, multiplie les démonstrations en la matière et augmente ses capacités balistiques. L'entrée de la Corée du Nord dans le club des pays nucléaires accroîtrait tous les dangers, mais toute tentative de dissuasion nécessiterait un cercle vertueux de paix et de désarmement mutuel.

la déclaration conjointe que viennent de publier les chefs d'État des cinq puissances nucléaires du Conseil de sécurité des Nations unies est un encouragement. On peut bien sûr la juger

Nous y voyons plutôt le résultat de la poussée en faveur du traité sur l'interdiction des armes nucléaires, que ces puissances ont certes refusé de signer au nom de leur attachement au TNP, mais qui a le mérite

Il faut aujourd'hui passer de la parole aux actes. Les urgences de la planète appellent le désarmement nucléaire. La péninsule coréenne n'est évidemment pas la seule concernée,

En 1950, après une série d'incidents et de fortes tensions à la frontière, la Corée du Nord envahit la Corée du Sud. Cette invasion déclenche une guerre par procuration entre les deux puissances nucléaires de l'époque, les États-Unis et la Chine, et provoque le premier grand bouleversement de la guerre froide. Celle que l'on appelle désormais la « guerre oubliée » fera environ un million de victimes militaires, deux millions de victimes civiles et de très nombreux disparus. Le 27 juillet 1953, la Corée du Nord, les États-Unis et la Chine signent un accord d'armistice. La Corée du Sud s'opposant au maintien de la partition en deux de la Corée n'a ni accepté l'armistice ni signé de traité de paix. C'est la raison pour laquelle, en dépit de la fin des combats, la guerre n'a diplomatiquement et officiellement jamais pris fin. Les espoirs de réconciliation ont brièvement été entretenus en 2000, puis de nouveau en 2018, avant de finalement tourner court. Aujourd'hui, États-Unis, Chine, Corée du Nord et Corée du Sud ont conjointement affiché leur volonté, sur le principe et sur une base théorique, de déclarer la fin de la guerre de Corée.

nécessaire dans une région du monde soumise à de nouveaux équilibres. Un tel accord permettrait notamment la création d'une véritable zone démilitarisée, des discussions sur la dénucléarisation ou la redéfinition de certaines frontières maritimes, qui restent floues par endroits. L'ancrage géographique des deux Corées les place au coeur de l'Indo-Pacifique, nouveau centre de gravité stratégique mondial. Et parce que les défis sécuritaires, économiques, technologiques et environnementaux qui sont aussi les nôtres, la France et l'Union européenne ont, dans cette région, des intérêts et des valeurs à défendre, et des partenariats à construire. La montée en puissance et les revendications territoriales de la Chine, exprimées de façon chaque fois plus appuyée, l'intensification de la compétition sino-américaine ou encore les tensions à la frontière sino-indienne modifient les équilibres régionaux. s'ajoutent des menaces transnationales persistantes, telles que la piraterie, le terrorisme, les trafics en tout genre, ainsi que les conséquences désastreuses du dérèglement climatique, dont les effets peuvent déjà se faire sentir en matière de sécurité. Toutes ces évolutions ont des répercussions directes sur l'ensemble de la zone, y compris sur les territoires français. La Corée du Sud et la France pourraient, dès lors, envisager de coopérer dans l'Indo-Pacifique en contribuant à apaiser les tensions dans la région et à maintenir un équilibre, tout en préservant leurs propres intérêts nationaux. Dans le contexte de récente redistribution des alliances dans la région- je pense en particulier à l'accord Aukus () -, la Corée du Sud et la France auraient intérêt à engager un dialogue en vue de coopérer dans l'Indo-Pacifique, ce qui permettrait d'accroître la confiance mutuelle et la convergence stratégique.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, guerre sans fin, orpheline de la guerre froide, l'interminable crise coréenne attire régulièrement l'attention de la communauté internationale.

de temps en temps, mais jamais complètement refermé. L'absence depuis 1953 d'un véritable traité de paix entre la République de Corée et la Corée du Nord est-elle propice à la poursuite des tensions ? Autrement dit, l'adoption d'une déclaration de la fin de la guerre de Corée serait-elle de nature à améliorer les choses ? À l'évidence, la réponse ne peut être que nuancée, compte tenu de la complexité d'une situation géopolitique sur laquelle plane encore aujourd'hui l'ombre des grandes puissances, les États-Unis, la Chine et la Russie. Hier comme aujourd'hui, celles-ci maintiennent sous différentes formes, y compris militaires, leur présence dans la zone. Si l'on ne peut ignorer les ambitions de grandeur de de la dynastie Kim pour son pays, force est aussi de constater que la péninsule reste un pion dans la région, comme elle l'a toujours été au cours du XX siècle. En effet, on connaît le principal ressort du déclenchement de la guerre en 1950 : la lutte pour la domination dans la région entre les L'enjeu a-t-il évolué depuis ? Si nous sommes heureusement sortis de la guerre froide, les luttes d'influence demeurent, ce qui n'est pas sans susciter des inquiétudes. Aujourd'hui, on le sait, les États-Unis ont déplacé leurs intérêts stratégiques vers la zone Asie-Pacifique. ses intérêts économiques, mais également à contenir la menace chinoise dans la région. Grâce au traité de défense conclu avec Séoul, la menace nord-coréenne offre une fenêtre stratégique au Pentagone pour surveiller la Chine. Dans ces conditions, dans le contexte d'un bras de fer stratégique, quel crédit accorder aux offres de pourparlers que l'administration Biden a faites l'été dernier au dirigeant nord-coréen ?

Depuis les jeux Olympiques d'hiver de 2018 en Corée du Sud, ce dialogue existe, mais il a produit peu d'effets à ce stade. Pour l'heure, en espérant que tous les acteurs impliqués prennent les engagements nécessaires à la mise en oeuvre d'un véritable dialogue,

Tout d'abord, nous le devons au peuple coréen. J'ajoute que nous le devons plus encore à celui du nord, qui, au-delà d'avoir en commun avec celui du sud la peur d'une escalade aux frontières du pays, doit en plus faire face à une situation économique très dégradée,

Aussi le texte de la proposition de résolution prend-il encore un peu plus de relief. En effet, la « dénucléarisation complète de la péninsule coréenne » doit être une préoccupation majeure de la communauté internationale. Enfin, mes chers collègues, la proposition de résolution s'inscrit tout simplement dans la tradition de défense de la paix et des droits de l'homme chère à la France. Fidèle à ses valeurs, notre pays ne peut se contenter, pour la péninsule coréenne, d'un simple et fragile cessez-le-feu. Le groupe RDSE votera donc cette proposition de résolution.

avec les deux Corées pour que ces pays puissent, selon les termes de la déclaration commune du 27 avril 2018, adopter une déclaration de la fin de la guerre de Corée et entamer un dialogue en vue de la signature d'un traité de paix. Le texte que nous examinons aujourd'hui enjoint également la France de soutenir les efforts internationaux en faveur d'une dénucléarisation complète de la péninsule coréenne.

Il est en effet urgent aujourd'hui de faire entendre la voix de la paix et du dialogue entre les deux Corées, en créant les conditions d'un véritable système de sécurité collective en Asie du Nord-Est, régions les plus militarisées du monde. Revenons sur les faits. Le 25 juin 1950, l'armée nord-coréenne franchit le 38 parallèle marquant la division de la péninsule entre le Nord et le Sud.

ont menacé le cessez-le-feu. Le Nord a placé à plusieurs reprises ses troupes en état de guerre. Malgré les tensions, les deux pays n'ont jamais complètement interrompu leur dialogue. Depuis des décennies, les deux Corées enchaînent des phases de confrontation et de rapprochement. En 2000 et 2007, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-il a tenu à Pyongyang deux sommets historiques avec les dirigeants du Sud.

ou empoisonnées par les velléités de Pyongyang de se doter de l'arme nucléaire et d'un arsenal balistique de longue portée, qu'il exhibe lors d'essais spectaculaires. Les États-Unis ont toujours fixé comme préalable à la fin de la guerre le renoncement par la Corée du Nord à son programme nucléaire militaire. Le nouveau président des États-Unis, Joe Biden, a fait le choix d'ignorer l'épouvantail nord-coréen pour se concentrer, autant que possible, sur sa priorité absolue : contenir la menace chinoise dans la sphère Asie-Pacifique. En marge de la reprise du dialogue avec les États-Unis, Kim Jong-un a renoué les liens avec la Chine, qui avaient pâti des purges de personnalités jugées trop pro-Pékin et de l'imposition des sanctions de

derrière ses frontières, surveillées par l'armée, qui a reçu l'ordre de tirer à vue sur toute personne essayant de passer. Officiellement, la Corée du Nord n'a enregistré aucun cas de covid-19. aucun cas de covid-19. Les experts en doutent, nous aussi. Les deux Corées ont multiplié les gestes d'apaisement au cours de l'année 2018, instaurant un climat de détente

Dans cette déclaration, les présidents sud et nord-coréens assuraient vouloir instaurer une paix durable et signer un traité de paix dans le courant de l'année. À cette occasion, les deux présidents ont également affirmé s'engager en faveur d'« une péninsule coréenne non nucléaire

de dénucléarisation, et à une réflexion sur la situation des familles séparées. Les enjeux diplomatiques sont

du président sortant, lequel ne peut se représenter. En revanche, ce qui est certain, c'est l'urgence, ressentie par la Corée, du Nord comme du Sud, de relancer le dialogue

s'achèvera en mars 2022. Quant à Kim Jong-un, il a surtout un besoin urgent d'aide pour faire face à la crise alimentaire qui s'aggrave dans son pays. Dans l'immédiat, la priorité pour la Corée du Nord est d'obtenir au plus vite une assistance alimentaire et médicale de la part de Séoul, afin de contrebalancer sa dépendance à l'égard de la Chine. Dans ces conditions, les deux pays auraient tout intérêt à mettre un terme à l'état de guerre qui les oppose depuis 1953.

protagoniste de la guerre de Corée, membre du Conseil de sécurité de l'ONU, n'est pas directement concernée par un tel traité de paix. Toutefois, elle exprime le souhait que les pourparlers à six, entre les deux Corées, les États-Unis, la Chine, la Russie et le Japon, reprennent. Alors que les tensions ne font que s'accroître dans la péninsule coréenne, l'adoption par la représentation nationale de la présente proposition permettrait

pour le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants. Monsieur

Le retour récent d'un transfuge nord-coréen- il était passé au sud -ayant réussi à pénétrer la Corée du Nord par la voie terrestre n'a pas manqué de nous rappeler que l'état de guerre est toujours en cours dans cette région du monde.

ces trois lettres symbolisent l'empêchement de la stabilité et de la paix dans la péninsule, déchirent bien des familles et hantent les Coréens, inquiets d'une possible reprise des hostilités, telle une épée de Damoclès. Dans ce contexte,

a présenté ses voeux pour la nouvelle année, le président Moon Jae-in a réaffirmé sa détermination à chercher une « voie irréversible vers la paix » et appelé à reprendre le dialogue et la coopération avec la Corée du Nord. On espérait donc, en raison de ces derniers développements, que l'année 2022 serait l'aube d'une nouvelle ère de paix et de prospérité, avec, enfin, une déclaration de fin de la guerre entre les deux Corées. Malheureusement, le lancement ce matin même par Pyongyang d'un projectile non identifié, qui pourrait être un missile balistique, a fait l'effet d'une douche froide. Ce nouvel essai survient en guise de réponse à la proposition de Washington, depuis l'arrivée au pouvoir du président Biden, de reprendre les négociations.

que l'on attendait des signes d'ouverture de la part de Kim Jong-un, son allocution devant le Parti du travail n'a nullement éclairé la communauté internationale sur ses intentions, ni sur les relations intercoréennes, ni même sur les négociations en matière de dénucléarisation avec les États-Unis. Il s'est contenté d'indiquer que, selon lui, « l'environnement militaire de plus en plus instable dans la péninsule coréenne et la situation internationale exigent le renforcement des capacités de défense nationale » du pays et la poursuite de son programme d'armement, sans mentionner Washington. Tout ceci est amèrement regrettable. Nous tenons à adresser une pensée toute particulière de solidarité aux habitants de la Corée du Nord, qui vivent aujourd'hui les dures conséquences de décennies de pénurie alimentaire.

ces questions sa priorité et qu'elle fasse un pas décisif vers la paix, la stabilité et la prospérité de la péninsule coréenne, pour le seul bénéfice de sa population. En dépit des derniers mauvais signaux, il est hors de question de baisser les bras. Compte tenu des tensions croissantes dans l'Indo-Pacifique, aboutir à la paix dans cette région constituerait un véritable espoir pour la paix et la stabilité mondiales. Nous formons donc le voeu

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis tentèrent d'endiguer la progression communiste partout où ils le pouvaient, la politique dite de . Occupée par les forces japonaises depuis le début du XX siècle, la Corée, libérée par les Alliés, a fait l'objet d'une partition Nord-Sud. En 1950, la Corée du Nord a tenté de remettre en cause ce partage et s'est lancée dans une offensive pour envahir la Corée du Sud. Sous l'égide de l'ONU, les États-Unis et leurs alliés sont alors venus au secours de Séoul. Les Soviétiques et les Chinois, quant à eux, ont soutenu Pyongyang. Après trois ans de guerre et plusieurs centaines de milliers de morts, le conflit s'est stabilisé autour de la ligne du 38 parallèle. La signature d'un armistice a sanctuarisé cette partition. Depuis près de soixante-dix ans, cette ligne divise la péninsule en deux, séparant des milliers de familles. la coexistence des deux Corées n'est guère pacifique. Ainsi, Christian Cambon nous a rappelé que la paix n'a jamais été signée. En 2006, la Corée du Nord a testé pour la première fois une arme nucléaire. Elle a procédé depuis à plusieurs essais nucléaires et balistiques, menaçant la sécurité de la péninsule et de toute la région. L'arme nucléaire sanctuarise le régime marxiste du Nord, qui entretient l'idée d'une menace d'invasion du Sud. C'est à cette condition que ce régime, d'un autre temps, parvient à se maintenir, tandis que sa population est opprimée. Le grand leader lui-même a reconnu récemment des tensions sur l'approvisionnement alimentaire et appelé ses compatriotes à se préparer à des temps difficiles. Nul doute que soixante-dix années de dictature les y auront bien préparés comme une épée de Damoclès sur la sécurité et la prospérité de la région. Tous les acteurs concernés ont intérêt à ce que les tensions prennent fin et que la péninsule coréenne cesse enfin d'être l'une des plus dangereuses poudrières de la planète.

président des États-Unis a cru, l'année suivante, pouvoir mettre un terme au conflit par la voie de la négociation. Le monde a suivi avec beaucoup d'attention la rencontre historique des deux chefs d'État en juin 2018. Les espoirs ont cependant été de courte durée, puisque la série des rencontres s'est achevée par celle de Hanoï

déjà significativement réduit les échanges internationaux. Que la Corée du Nord se referme sur elle-même n'est pas une bonne nouvelle pour la paix. Notre vieux continent européen a réussi depuis la fin du dernier conflit mondial à tenir en respect le spectre de la guerre. Nous sommes persuadés que la préservation de la paix en Europe

Montesquieu, « l'effet naturel du commerce est de porter à la paix. Deux nations qui négocient ensemble se rendent réciproquement dépendantes : si l'une a intérêt d'acheter, l'autre a intérêt de vendre ; et toutes les unions sont fondées sur des besoins mutuels. » La construction de l'Union européenne prouve l'efficacité de ces principes, et ce depuis le début de la guerre de Corée. La proposition de résolution de Christian Cambon nous engage à oeuvrer pour la paix entre les deux Corées. Je salue cette initiative, soutenue par la Corée du Sud, en espérant que les assemblées des États-Unis,

Merci

de la France dans cette région, qui s'est traduite par l'engagement et le sacrifice des soldats français volontaires dans le bataillon français de l'ONU. Nous devons honorer leur mémoire et continuer à jouer un rôle dans cette zone en participant à l'établissement d'une paix durable.

La deuxième raison a trait à l'actualité géopolitique. En dépit de la fin des hostilités, le 27 juillet 1953, la péninsule coréenne ne bénéficie pas d'une paix pleine et entière. La stabilité relative des relations entre la République populaire démocratique de Corée et la Corée du Sud repose sur une convention d'armistice signée par les commandants des trois parties aux négociations de paix celui des forces des Nations unies, celui de l'Armée populaire de la République démocratique de Corée, devenue Corée du Nord, et celui de l'Armée des volontaires du peuple chinois. Or le regain des tensions et les démonstrations de puissance récurrentes des États de la région fragilisent fortement un processus de paix inachevé. Ne serait-il pas temps de trouver un prolongement à un armistice qui dure depuis près de

armes nucléaires (TNP). Sa « sortie » du TNP et la poursuite de son programme militaire, accompagnée de plusieurs essais, ont contribué à une escalade des plus dangereuses pour la sécurité mondiale. Cependant, l'histoire a- tragiquement ! - démontré les limites de la politique d'isolement diplomatique des nations. Aussi semble-t-il opportun que la France puisse, d'une part,

Alors que la France exerce la présidence de l'Union européenne, son implication pourrait favoriser une mobilisation plus large et une concertation fondée sur le renouveau. C'est aussi, à mon sens, l'occasion de faire la démonstration de la singularité française, respectueuse de toutes les parties et du multilatéralisme.

constituent des leviers indispensables pour créer les conditions d'une paix pérenne. Cette proposition de résolution invite le Gouvernement à y ajouter un volet supplémentaire, le volet diplomatique. Enfin, mes chers collègues, au-delà des États et des armes, il y a des êtres humains, des générations au Nord et au Sud qui méritent que nous nous mobilisions pour la paix. La parole

soixante-dix ans n'offre pas un cadre stable aux relations entre les deux Corées et les pays parties à la guerre de Corée. La France a tout intérêt à soutenir les initiatives en faveur de l'adoption d'une déclaration de fin de la guerre, gage de stabilité dans une région stratégique. Lors de la dernière visite d'État du président sud-coréen Moon

sur les grandes questions internationales ; le développement de la coopération en matière de diplomatie, de sécurité et de défense ; l'approfondissement des relations économiques le développement des échanges et de la coopération dans les domaines des sciences, de l'enseignement, de la culture et des sports. Ces principes ont été réaffirmés lors du dialogue stratégique qui s'est déroulé en mai 2019 entre les ministres des affaires étrangères français et coréen. L'adoption d'une déclaration de fin de la guerre permettrait également d'aborder la question de la dénucléarisation de la péninsule coréenne, condition d'une paix pérenne. En effet, si la si la question du nucléaire chinois prend de l'ampleur, compte tenu des diverses avancées technologiques de la Chine, celle du nucléaire nord-coréen reste préoccupante. La détente relative que Donald Trump et Kim Jong-un avaient tenté d'instaurer après leur première rencontre à Singapour, en juin 2018, n'a en effet pas permis de faire avancer le dossier de la dénucléarisation dans la région. La Corée du Nord n'a certes pas réalisé de nouveaux essais nucléaires depuis septembre 2017, mais elle a testé à plusieurs reprises le lancement d'engins susceptibles de transporter des ogives nucléarisées.

la Corée du Nord continuait de faire progresser ses programmes d'armement nucléaire et de missiles malgré les sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et les efforts diplomatiques de haut niveau,

Enfin, en août dernier, l'Agence internationale de l'énergie atomique indiquait que les Nord-Coréens avaient relancé leur réacteur nucléaire de Yongbyon,

appelle le Gouvernement à oeuvrer à l'adoption d'une déclaration de la fin de la guerre de Corée, est une bonne initiative, dont l'exécutif apprécie l'esprit et la méthode.

durant les combats meurtriers qui se sont déroulés entre 1950 et 1953, en particulier lors de la bataille de Crèvecoeur à l'automne 1951.

poursuivi ces derniers mois le développement de ses programmes nucléaire et balistique, en violation des résolutions du Conseil de sécurité. Dans le domaine nucléaire, le dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique, publié en août dernier, fait état d'une reprise, après plusieurs années d'arrêt, de l'activité des installations de Yongbyon. Il s'agit du principal site nucléaire du pays, où se situe s'agit du principal site nucléaire du pays, où se situe un réacteur permettant de produire du plutonium de qualité militaire. En parallèle, la Corée du Nord a effectué en septembre et en octobre 2021- il y a donc très peu de temps -cinq séries de tirs de missiles, toutes préoccupantes, mais dont deux attirent plus particulièrement notre attention. Le 28 septembre dernier, quelques jours après une nouvelle proposition de déclaration de la fin de la guerre de Corée par le président Moon Jae-in, lors de la 76 session de l'Assemblée générale des Nations unies, le régime nord-coréen a annoncé avoir réussi un test de tir de missile intégrant un planeur hypersonique, qui constitue une nouvelle génération de missile dont seul un nombre très restreint d'États disposent aujourd'hui. Le 19 octobre, la Corée du Nord

En posant les jalons d'un renforcement significatif et continu des forces nucléaires nord-coréennes, cette séquence a confirmé la priorité que continue d'accorder le régime à l'amélioration et au

: les autorités sud-coréennes et japonaises viennent d'annoncer un nouveau tir de projectile effectué par la Corée du Nord, qui semble s'apparenter à un tir de missile balistique. Au moment où je vous parle, des vérifications sont en cours pour en déterminer la nature exacte. En tout cas, face à une telle attitude, nous sommes tous mobilisés autour d'un objectif très clair : le retour rapide, et en toute bonne foi, de la Corée du Nord à la table des négociations, lesquelles sont destinées à obtenir la dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible du pays, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité. J'y insiste : dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible ! À ce titre, la mise en oeuvre par l'ensemble de la communauté internationale de l'ensemble des sanctions décidées par le Conseil de sécurité demeure aujourd'hui, faute de mieux, l'instrument fondamental dont nous disposons pour lutter contre la prolifération nucléaire et balistique nord-coréenne.

maintenant à la proposition de résolution. Ce texte se rapporte à une initiative que le président de la République de Corée, M. Moon Jae-in, a prise en septembre dernier devant l'Assemblée générale des Nations unies,

l'a fait savoir lors d'échanges avec le président Moon Jae-in, la France est favorable à toute initiative visant à apaiser les tensions dans la péninsule coréenne, dans le respect des résolutions du Conseil de sécurité.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, il est des moments dans la vie d'un élu où l'on peut ressentir une légitime fierté pour le travail que l'on a accompli. Tel est bien le sentiment que je souhaite partager avec vous en cet instant. Le Sénat, une fois de plus,

Il est tout d'abord nécessaire de rappeler que la loi du 17 mai 2011 a substitué à la réglementation nationale en matière de défense extérieure contre l'incendie le principe d'une réglementation départementale, départementale, établie par le préfet en concertation avec les élus locaux, l'objectif étant de répondre aux spécificités des différents territoires. Dix ans après l'adoption de cette loi, force est de constater que cette réforme, souhaitée par les élus, notamment par l'Association des maires de France, n'a pas répondu à leurs attentes. Elle a, au contraire, provoqué un large mécontentement des maires,

Selon l'enquête que nous avons menée, 70 % des maires considèrent que la concertation n'a pas été satisfaisante, et 81 % d'entre eux estiment que leur territoire n'est que partiellement couvert au regard des nouvelles normes.

Cette situation conduit de nombreux maires à refuser toute autorisation d'urbanisme, enclenchant ainsi un cercle vicieux de baisse de population- et donc de ressources -et de fermeture des classes. À l'heure où la revitalisation des territoires ruraux s'impose comme une priorité et où des crédits importants sont consacrés à cet objectif, les règlements départementaux de défense extérieure contre l'incendie (RDDECI) viennent trop souvent nuire aux actions menées en ce domaine.

selon nous, complété par un audit national de la DECI conduit par l'État. Cette recommandation a d'ailleurs été accueillie favorablement par le ministre de l'intérieur lorsque nous lui avons présenté notre rapport le 7 décembre dernier.

Il nous paraît aussi nécessaire de faire précéder les décisions relatives au règlement départemental d'une étude d'impact, afin de mesurer les conséquences financières de ces décisions sur les communes et de mieux prendre en compte les autres solutions possibles. Je pense par exemple aux bâches et autres points d'eau naturels pouvant être utilisés dans un cadre contractuel maîtrisé- cela renvoie d'ailleurs à la problématique plus générale de l'eau en milieu rural. Il faut en outre insister sur la nécessité d'une méthodologie de concertation, exigeante et précise, des acteurs de la défense extérieure contre l'incendie. Jusqu'à présent, la concertation a trop souvent été plus formelle que réelle. Le périmètre des acteurs concernés comprend certes les partenaires institutionnels et les organisations d'élus, mais il doit s'élargir à l'ensemble des maires. L'une des principales barrières à la mise en conformité des communes, en particulier les plus petites d'entre elles dans les zones rurales, est son coût. C'est pourquoi un soutien budgétaire significatif de l'État s'impose.

La dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) pourrait également être davantage mobilisée. Actuellement, ce n'est pas le cas dans tous les départements. Le recours à cette dotation devrait être généralisé dans chaque département, pour des montants pouvant aller jusqu'à 100 % du coût du projet à financer, en fonction de critères à définir avec les maires. Après avoir ainsi répondu à l'urgence, il sera nécessaire de faire un bilan, dans trois ans, de cette mobilisation accrue de la DETR et du financement par le plan France Relance, et de réfléchir à une source de financement plus pérenne. pérenne. Les normes en matière de défense extérieure contre l'incendie doivent désormais être figées, et ce après avoir intégré les moyens des SDIS dans les arbitrages à rendre. Il faut en effet choisir des solutions garantissant une répartition optimale des coûts entre les SDIS et les communes.

En France, la culture du risque est peu répandue et inégalement diffusée. Il est surprenant que l'obligation d'installation d'un détecteur de fumée, effective depuis 2015, soit si peu respectée et qu'elle ne fasse que très rarement, voire jamais, l'objet d'un rappel. Le renforcement de l'autoprotection doit favoriser, en retour, l'assouplissement des règles imposées aux communes. Enfin, dans cette approche rénovée, le numérique et les innovations technologiques offrent des pistes intéressantes d'optimisation de la défense contre

nous devons rechercher cet équilibre entre les moyens mobiles des SDIS et les ressources communales. Le référentiel national de la DECI se contente de fournir un cadre méthodologique,

en lui consacrant une mission d'information. J'adresse toutes mes félicitations à ses rapporteurs, Hervé Maurey et Franck Montaugé, pour le travail qu'ils ont réalisé. Les représentants des territoires que nous sommes savons à quel point ce sujet est important et sensible localement. Celui-ci me tient particulièrement à coeur, non seulement en tant qu'élu local, mais aussi en tant qu'ancien colonel de sapeurs-pompiers professionnels.

Pour la plupart des communes rurales, où le bâti est diffus et l'habitat morcelé, les obligations imposées par les règlements départementaux de DECI sont très souvent source d'insatisfaction, compte tenu des contraintes urbanistiques, financières et juridiques

d'État, quelles consignes le Gouvernement entend-il donner aux préfets pour que la loi de 2011 soit respectée et que les règlements départementaux ne soient pas la copie conforme du règlement national, mais bien le reflet d'une prise en compte des réalités de terrain que vous venez d'évoquer ?

et de porter une appréciation sur cette politique à l'échelle de leur territoire, par manque de compétences techniques. Il y a donc, d'un côté, la complexité des règles qui vient empêcher, presque de fait, une appréciation décentralisée de la DECI par les élus locaux et, de l'autre, la rigidité du cadre normatif qui vient bloquer fondamentalement toute démarche de différenciation. il faudrait ajouter les difficultés budgétaires qu'occasionne ce service dans les territoires ruraux. Face à toutes ces contraintes qui tiennent les élus locaux en échec, il existe un régime de responsabilité particulièrement exigeant, parfois confus, mêlant responsabilité administrative de la commune et responsabilité personnelle du maire. Chacun sait que, depuis les années 1990, le juge administratif a cessé de requérir une faute lourde pour engager la responsabilité administrative d'une autorité publique. Cela vaut pour l'autorité communale en cas de sinistre lié à la défaillance des services de lutte contre l'incendie. Nos administrations locales font donc face à un régime particulièrement pointilleux, quand bien même, comme l'a souligné le rapporteur public Vincent Villette dans ses conclusions sur l'arrêt rendu par le Conseil d'État le 18

Pour ma part, je voudrais revenir sur la question du volontariat. Le manque d'effectifs de sapeurs-pompiers volontaires est réel et pose un véritable problème dans de nombreux départements. Le Parlement a adopté à l'automne la proposition de loi, dite Matras,

Cette bonification a été remplacée par un renforcement de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance (NPFR). Or la revalorisation des montants de cette prestation n'est prévue que par voie réglementaire.

Il est urgent d'aboutir à un dispositif progressif permettant de fidéliser et de récompenser les sapeurs-pompiers volontaires. Je vous rappelle à ce sujet que, devant le congrès de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, qui s'est tenu à Marseille, le Président de la République a indiqué vouloir reprendre l'idée d'une bonification de la retraite

en novembre dernier, le Président de la République a annoncé une revalorisation de cette prestation, dont le financement- vous le savez tous très bien ici -est partagé entre les SDIS et l'État. Un travail est donc en cours, en lien avec les financeurs des SDIS, pour définir

Messieurs les rapporteurs, vous préconisez à ce titre de « faire émerger une " culture du risque " », notamment en sensibilisant les populations au risque d'incendie. Je partage entièrement cet objectif, mais je m'interroge sur la mise en oeuvre concrète de votre proposition. Comment lutter contre la multiplication des incendies, alors

qui pourrait bien se révéler très utile, à travers la création de réserves citoyennes des services d'incendie et de secours, ouvertes aux citoyens de plus de seize ans. Concrètement, dans quelle mesure ces réserves citoyennes peuvent-elles contribuer à faire émerger une culture du risque en France ? comment le Gouvernement compte-t-il suivre la mise en place des réserves citoyennes, qu'il s'agisse des missions qui leur seront confiées ou de leur organisation ? Ces réserves pourraient, je le crois, devenir des relais indispensables dans la prévention et la lutte contre les incendies,

La réforme de 2011 semble ne pas avoir véritablement répondu aux attentes des élus ruraux, qui regrettent que cette transformation de la politique de défense incendie n'ait pas apporté une réponse mieux adaptée à la réalité des territoires. Le coût de la mise aux normes de la défense incendie a souvent dépassé la capacité financière de nombreuses petites communes rurales, les obligeant à renoncer à des projets d'investissement futurs, faute de ressources suffisantes. En effet, le coût de l'installation des bornes d'incendie ou celui de la révision des réseaux d'eau représente une somme considérable pour de modestes budgets communaux. De même, l'obligation d'une distance maximale entre les points de raccordement au réseau d'eau et les habitations porte atteinte à l'attractivité des petites communes. Désormais, toute nouvelle construction doit se situer à moins de 200 mètres d'une borne incendie, cette distance étant portée à 400 mètres si l'habitation est isolée. Cette contrainte nuit à la capacité des communes à délivrer des permis de construire. Elle entrave ainsi l'installation de nouveaux habitants, indispensable au dynamisme, voire à la survie de ces territoires, au moment même où ceux-ci retrouvent une vraie attractivité. Progressivement, les élus se sont aperçus que la mise en conformité avec les normes de défense incendie constituait une entrave au développement et à la revitalisation des territoires ruraux. Il apparaît donc primordial d'accompagner les communes dans cet effort. Pourquoi, madame la secrétaire d'État, ne pas créer ou recréer des retenues collinaires dans les endroits les plus isolés ? Une des préconisations des rapporteurs consiste à affecter 1,2 milliard d'euros sur trois ans

par rapport aux risques et entraîner des coûts de mise aux normes très importants pour les budgets des communes rurales, constitue un sujet prégnant dans nos territoires. Ainsi, quand la commune ne dispose pas de terrains, elle doit acquérir du foncier pour l'installation des bâches, dont la durée de vie excède à peine Si un accompagnement financier permettant d'alléger la facture est possible la dotation d'équipement des territoires ruraux, la DETR, ou l'aide des conseils départementaux, il n'en demeure pas moins que, pour certaines communes, la mise en conformité prendra plusieurs années, au détriment de projets structurants. Quelles seront en outre les conséquences en termes de responsabilité des maires en cas d'incendie d'une construction dans une zone ne répondant pas aux caractéristiques du règlement départemental ? À titre d'exemple, en Charente-Maritime, pour une intercommunalité regroupant 129 communes, 25 millions d'euros sont nécessaires pour l'installation de 2 500 bâches. Des projets d'urbanisme sont bloqués en raison d'une règle qui impose une distance minimale entre le point d'eau et l'habitation, obérant la dynamique de nos territoires ruraux. Dans leurs conclusions, les rapporteurs, que je salue, regrettent que la réforme de la DECI n'ait pas tenu ses promesses, et qu'elle ait engendré des obligations accrues et inadaptées aux réalités locales, avec des conséquences fâcheuses sur l'attractivité et le développement des communes rurales.

au même stade ... Ma question sera simple, madame la secrétaire d'État : quand allez-vous solliciter les préfets pour démarrer cette évaluation préalable indispensable à la révision des règlements départementaux ? Quant aux préfets, ils appliquent tout simplement les règlements départementaux ; ils attendent donc votre impulsion

mais il a aussi modifié les règles de contrôle des points d'eau. Désormais, seuls les points d'eau naturels et artificiels restent de la compétence des SDIS, du fait de la nécessité de disposer de pompes qu'eux seuls sont en capacité de déployer. En revanche, il revient aux communes de contrôler les poteaux et bouches d'incendie.

ou, en cas de transfert de cette compétence, de celle du président de l'EPCI. Ce pouvoir de police spéciale vient compléter le pouvoir de police générale du maire en matière de prévention et de lutte contre les incendies.

Si les enjeux sont techniques, tout le monde est capable de saisir les contraintes de fond : d'une part, assurer la sécurité des personnes et des biens, en adéquation, bien sûr, avec les normes en vigueur ; d'autre part, disposer de moyens humains, techniques et financiers à mobiliser.

s'agit de rechercher par le dialogue un consensus qui s'avère nécessaire et de sortir ainsi de l'arbitraire et de la dictature des normes. Il s'agit aussi de partager et de diffuser une culture du risque et, peut-être, de ses conséquences,

des critères de différenciation permettant une déclinaison encore plus adaptée aux spécificités locales ? La parole est

n'ose imaginer quelle aurait été votre réaction si nous avions suivi la démarche inverse en renforçant le dispositif descendant

donner aux élus locaux, qui sont dans l'impossibilité de mettre en oeuvre ce grand principe du code

De fait, un soutien budgétaire de l'État s'impose, en particulier pour les collectivités les plus petites et les plus fragiles financièrement.

ou de la consultation des élus. Le rapport très fouillé de nos collègues Hervé Maurey et Franck Montaugé se fait l'écho des préoccupations de nombreux élus ruraux. estiment que leur voix ne porte pas assez dans la concrétisation de cette politique cruciale. Pourtant, c'est précisément la problématique des zones rurales qui a justifié, en 2009, le premier encadrement législatif de la DECI. L'article 6 du règlement national prévoit bien la consultation des « acteurs concernés » en amont de l'élaboration du règlement départemental. Malheureusement, le périmètre retenu varie dans les faits d'un département à l'autre.

le cas d'une commune qui avait sollicité le soutien financier de l'État pour l'installation de points d'eau. Le département avait été conduit à relayer cette demande. De semblables démarches pourraient être, sinon évitées, du moins anticipées, par une plus large

Vous le comprendrez aisément : nos inquiétudes demeurent, car la mandature actuelle s'est jusqu'ici révélée décevante pour nos collectivités. La parole est à Mme Agnès Canayer.

je m'en tiendrai aux seuls problèmes de la concertation avec les élus et de l'élaboration du schéma communal ou intercommunal de DECI.

énonce vingt propositions pertinentes, qui, autour de cinq axes, visent à parvenir à une défense extérieure contre l'incendie équilibrée et proportionnée. plus particulièrement sur l'accompagnement des communes et les possibles financements des schémas communaux ou intercommunaux permettant de trouver des solutions locales adaptées pour améliorer la DECI.

préconisent la création d'une ressource complémentaire pour permettre aux communes de réaliser ces investissements sans mobiliser de manière excessive la DETR.